... Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. L'ordre du jour appelle la désignation des membres de trois commissions spéciales chargées d'examiner le projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, le projet de loi portant suppression de surtranspositions des directives européennes en droit français et le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, En application de l'article 8, alinéas 3 à 11, et de l'article 10 de notre règlement, les listes des candidats établies par les groupes ont été publiées. Elles seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure.

une « start-up judiciaire », un tribunal de grande instance qui recevrait toutes les demandes d'injonction de payer. L'injonction de payer est une procédure qui existe depuis fort longtemps. Elle permet à un créancier d'obtenir un titre qui devient exécutoire s'il n'y a pas d'opposition et de recouvrer une créance. Pour simplifier, on peut dire qu'elle est essentiellement utilisée par les organismes de crédit et, éventuellement, par des propriétaires pour recouvrer des loyers.

ne traiter que des dossiers et ne jamais recevoir de justiciables. La commission a accepté votre proposition à peine modifiée, ce qui, je l'avoue, m'a laissé très perplexe. Nous avons déposé un amendement de suppression

Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure technique pour répondre à l'attente du justiciable, sauf à vouloir faire plaisir aux créanciers institutionnels

Rappelons que le droit à un recours effectif est garanti par l'article XVI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le droit à un procès équitable par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés son effectivité sera dérisoire compte tenu notamment de la dématérialisation imposée, du flou sur la juridiction compétente, de l'éloignement géographique de la juridiction nationale et, bien sûr, de la vulnérabilité de la plupart des personnes concernées. En effet, rien n'assure que la personne visée par l'injonction de payer sera en capacité d'accéder à internet ou d'y exercer correctement ses droits. Dans son dernier rapport d'activité, le Défenseur des droits estime que 27 % des personnes ne peuvent utiliser ou ne maîtrisent pas l'outil informatique, sans compter les personnes qui maîtrisent l'outil, mais ne maîtrisent ni le droit ni la procédure civile et ne seront pas en capacité d'exercer seules un recours. Ainsi, la dématérialisation constitue à n'en pas douter un obstacle à l'accès au juge et à l'effectivité du recours. De manière plus générale, nous nous opposons à la dématérialisation intégrale des petits litiges, car ce sont précisément ces contentieux qui nécessitent une comparution physique, notamment pour la mise en oeuvre de la procédure orale- qualification par le juge des demandes, tentative de conciliation, office de protection du juge en matière d'intérêts des parties en situation de dépendance ou de domination. En outre, et comme le souligne d'ailleurs le Syndicat de la magistrature, nous ne pouvons tolérer davantage la condescendance qui conduit à traiter ces contentieux avec légèreté au motif qu'il s'agirait de « petits » litiges. Rappelons qu'une somme

le remboursement d'un prêt, un conflit de loyer, une dette de 500 euros ... Ces petits litiges, parfaitement traités aujourd'hui par les juges d'instance, le seront demain par un tribunal " virtuel

ne doit pas se traduire par une justice expéditive au préjudice de l'humain et des plus vulnérables, particulièrement des plus pauvres. Quel est l'avis de la commission ? Le

le corapporteur indique qu'une souplesse a été intégrée par la commission, ce qui est exact, car désormais le recours à la procédure dématérialisée n'est plus une obligation, mais une possibilité. Il faut toutefois

qui sera compétente pour les injonctions de payer, dont on devine, car ce n'est pas explicite dans le texte, qu'elle sera également compétente dès lors que l'opposition ne porterait que sur des délais de paiement,

avec ce tribunal spécial, avec cette « start-up judiciaire » un système de traitement informatisé. Ils auront les réponses, et ils gouverneront le recouvrement de créances ! Voilà vers quoi vous nous conduisez, mais il est vrai que

c'est seulement au stade de l'ordonnance d'injonction de payer qu'une notification est adressée au débiteur, et c'est à ce moment-là qu'il est informé qu'une procédure a été intentée contre lui. Le débiteur

en ce qui concerne le fonctionnement et la protection des données, parce que, chaque fois que l'on numérise et que l'on centralise un dispositif, cela comporte un risque pour les procédures et pour les justiciables.

Il vise tout d'abord à exclure de la compétence du tribunal de grande instance spécialement désigné le traitement des requêtes en injonction de payer qui relèvent de la compétence des tribunaux de commerce. Nous souhaitons ainsi ainsi apporter une précision terminologique de nature à assurer le respect de la compétence matérielle des juridictions commerciales. Les requêtes en injonction de payer qui sont traitées par la juridiction spécialement désignée ne comprendront pas celles relevant des tribunaux de commerce. En revanche, les requêtes qui relèvent des tribunaux mixtes de commerce ou de la chambre commerciale en Alsace-Moselle seront traitées par la juridiction unique dématérialisée. Tel est l'objet du premier point de cet amendement. point de cet amendement. Le présent amendement vise ensuite à rendre obligatoire la saisine par voie dématérialisée du tribunal de grande instance spécialement désigné. La commission des lois avait souhaité introduire un peu plus de souplesse dans la forme de la saisine de la juridiction. Il nous semble toutefois important d'assurer un traitement dématérialisé qui sera sans doute plus efficace pour des créances d'un montant déterminé et qui résultent d'un contrat ou d'une obligation statutaire. La saisine dématérialisée permettra en effet de constituer un dossier unique et structuré, notamment dans des contentieux de masse tels que celui des crédits à la consommation, pour lesquels les pièces sont très nombreuses. Il nous semble que la dématérialisation permettra dans ce cas d'assurer un traitement plus rapide

Il sera également possible d'adresser au service d'accueil unique du justiciable des demandes d'aide pour que les personnes puissent réellement mettre en place cette saisine dématérialisée. L'accès au juge et l'égalité de traitement seront ainsi préservés.

la commission ? Le présent amendement du Gouvernement tend à préciser que la juridiction nationale des injonctions de payer ne traitera pas des injonctions relevant de la compétence du tribunal de commerce. Cette précision nous semble utile, comme nous l'avons d'ailleurs mentionné dans le rapport. En revanche, le rétablissement de la saisine dématérialisée comme seule voie d'accès ne nous semble pas acceptable. Elle est contraire à la position de la commission. En conséquence, je demande que l'amendement soit mis aux voix par division, en application de l'article 42,

de délais de paiement auprès d'un unique tribunal, solution qui pourrait permettre de réduire utilement les délais de traitement. En revanche, il nous paraît nécessaire de préserver l'accès à la justice de nos concitoyens et de leur laisser la possibilité de former leur recours physiquement dans le tribunal le plus proche de leur lieu de résidence. Cet accueil physique est de nature à rassurer les personnes les plus vulnérables, à charge ensuite pour ce tribunal de faire suivre la requête au tribunal compétent.

ou le tribunal d'instance. La commission ayant approuvé le principe de cette nouvelle juridiction, en y apportant des garanties, elle émet, sur cet

? Cet amendement tend à supprimer la possibilité de former opposition aux ordonnances par voie dématérialisée, au motif que celle-ci ferait intervenir un algorithme. Or ce n'est pas du tout le cas, puisque le règlement général sur la protection des données personnelles ne le permet pas.

régissant les procédures en la forme des référés devant les juridictions judiciaires, afin d'unifier et d'harmoniser le traitement des procédures au fond à bref délai. Pour être brève, je dirai l'objectif comptable d'un tel dispositif au final est à peine voilé, ce qui pose encore plus problème étant donné le véhicule légal choisi, la voie réglementaire, par l'intermédiaire d'une ordonnance. Les mesures réglementaires qui seront prises par le Gouvernement semblent préparer une future réforme de la procédure civile, notamment avec la création d'un acte unifié. En proposant de supprimer cet article, nous alertons sur les dispositions qui seront adoptées par voie réglementaire en matière de procédure civile, donc de droit privé. Celles-ci pourraient, pour une bonne part, être bien plus importantes et avoir un impact bien plus significatif que les dispositions qui nous sont proposées par voie législative, au travers du présent projet de loi. J'oserai dire que c'est une méthode chère au Président de la République, une méthode bien rodée, notamment depuis la loi Macron.

J'appelle aussi votre attention sur le fait que cette procédure s'applique dans différentes hypothèses en dehors de celle du référé, puisque le code de procédure civile vise parfois les décisions prises « en la forme des référés » des référés » ou « comme en matière de référé ». L'étude d'impact du projet de loi, que nous avons lue avec intérêt, madame la ministre, précise que treize codes ainsi que six lois prévoient, dans leurs dispositions législatives, le recours à cette procédure, avec des appellations très diverses : des procédures « en la forme », « selon la forme », « dans la forme », « comme en la forme », « sous la forme » et « comme en matière

Vous avez raison, monsieur le sénateur Sueur : en principe, nous sommes dans le domaine de la procédure civile, qui relève du pouvoir réglementaire. Toutefois, le législateur est intervenu à plusieurs reprises

Mais, dans les cas les plus complexes- par exemple, quand le patrimoine l'exige -, ce contrôle sera effectué par des professionnels, et non plus par les directeurs de greffe. Au fond, nous ferons appel à une véritable expertise

Toutefois, la commission préfère le dispositif gradué qu'elle a adopté s'agissant de la transmission de l'inventaire au juge, avec un délai supplémentaire, si celui-ci est justifié,

permettant de maintenir un contrôle par défaut du greffe, sous le contrôle du juge en cas de difficulté, tout en modernisant le système, alors que le dispositif du Gouvernement reviendrait à une

explication de vote. La commission des lois a choisi de maintenir le droit en vigueur s'agissant de la dispense d'établissement et de contrôle des comptes de gestion, qui peut être autorisée par le juge des tutelles en cas de modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée. En effet, il n'y a aucune raison d'élargir la possibilité de dispense aux mesures de protection confiées aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Le rapport de la mission interministérielle confiée à Mme Anne Caron-Déglise fait d'ailleurs état du souhait des membres de cette mission que les comptes établis par les mandataires professionnels

à la force publique en matière familiale. En effet, la commission a fait le choix de supprimer, dans le dispositif d'exécution des décisions en matière familiale que je vous propose, la possibilité pour le procureur de la République d'utiliser directement la force publique.

sont évidemment extrêmement douloureuses. Bien sûr, mes services peuvent inviter ces parents à porter plainte pour non-représentation d'enfant, mais cette voie pénale ne permet absolument pas l'exécution de la décision. Ainsi, au plan civil, le parent qui est confronté à un tel refus doit de nouveau saisir le juge aux affaires familiales pour solliciter la modification des dispositions non respectées, voire le changement de résidence habituelle de l'enfant. Cela n'est pas satisfaisant.

Bien évidemment, ce mécanisme ne peut reposer sur un recours systématique à la force publique et à l'exécution forcée. C'est pourquoi il est proposé un système gradué, qui permettra le prononcé d'amendes civiles et d'une médiation, y compris post-sentencielle. Toutefois, en dernier recours, lorsque ni la menace ni le prononcé d'une sanction financière, d'une part, ni la médiation, d'autre part, n'auront permis l'exécution spontanée de la décision rendue en matière de responsabilité parentale, la force publique doit pouvoir être utilisée. Il est donc proposé que le recours à la force publique soit requis par le parquet directement dans les cas les plus extrêmes. Je souhaite souligner qu'il existe déjà des modes d'exécution forcée en matière familiale. Le code civil prévoit déjà que le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.

qui me semble souhaitable et pertinente dans certaines situations et qui permet à l'ensemble du dispositif progressif que j'ai évoqué d'être dissuasif, et donc d'être respecté.

Soilihi, pour présenter l'amendement n° 241. L'article 18 du projet de loi vise à doter le juge aux affaires familiales d'un éventail d'outils lui permettant de rendre plus effective l'exécution des décisions prises en matière d'exercice de l'autorité parentale. Cet amendement vise à revenir sur la position de la commission, qui a supprimé la possibilité d'avoir recours à la force publique pour faire exécuter une décision relative à l'exercice de l'autorité parentale.

: le recours à la force publique doit être réservé aux cas les plus extrêmes. Il est important que cette ultime étape puisse être utilisée en dernier recours. Cela dit, je retire mon amendement.

n° 221. En effet, nous avons souhaité supprimer la possibilité de saisir sans condition le procureur de la République pour qu'il requière le concours de la force publique afin de faire exécuter les décisions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale. parentale. Selon le Gouvernement, cette procédure serait conçue comme une voie d'exécution ultime, réservée à certaines situations seulement- on imagine qu'il s'agit des situations les plus délicates. dans la rédaction qui est proposée, il n'y a pas de limite à l'application de cette procédure aux cas les plus graves ou aux hypothèses de refus réitérés Certes, il reviendra aux parquets de juger de l'opportunité de requérir la force publique- nous en sommes conscients -, mais ce ne sera pas neutre en termes d'alourdissement de la charge de travail des procureurs de la République : dès lors que la décision ou la convention ne sera pas exécutée, le juge mais la convention ne sera pas exécutée, le juge mais aussi la personne intéressée pourront saisir directement le procureur de la République, sans qu'aucune condition limite

vise lui aussi à rétablir la possibilité pour une personne directement intéressée ou pour le juge aux affaires familiales de saisir le procureur de la République pour qu'il requière le concours de la force publique, mais, cette

pour autant déclencher ce pouvoir- qui est un peu l'arme atomique -dans des conditions qui ne seraient pas justifiées d'un point de vue strictement humain. Nous devons penser avant tout à l'intérêt des enfants arrachés

sur ces différents aspects nous ont conduits à ne pas rejeter en bloc la proposition du Gouvernement, mais à essayer de la rendre praticable sans porter préjudice, par une

Monsieur le président Bas, vous avez bien lu notre texte, mais peut-être pas encore assez bien, puisqu'il est écrit que le procureur de Comme dans toutes les situations identiques, les démarches préalables au recours à la force publique seront fixées par décret. Elles le seront, comme elles le sont quand il est fait recours à la force publique pour l'exécution de

pourra éventuellement avoir recours à la force publique. On pourrait ainsi envisager qu'un huissier soit en charge d'une sommation. Ce précédent qui est efficace dans les situations à caractère international, telles que celles que j'évoquais, constitue un exemple dont le Gouvernement pourrait s'inspirer dans le contexte En toute hypothèse, il ne nous paraît pas opportun d'exiger une démarche préalable auprès d'un OPJ. C'est pourquoi je ne suis pas favorable à l'amendement de Mme la sénatrice Muriel

Madame la ministre, je comprends ce que vous recherchez. Vous avez probablement sur votre bureau de nombreux dossiers, pas tous identiques, concernant des questions de non-représentation d'enfant, qui sont souvent des situations extrêmement dramatiques. Cela étant, dans ces dossiers, l'idée qu'il faudrait permettre à la force publique d'intervenir pour appliquer une décision du juge aux affaires familiales

d'obtenir des juges, parce qu'il n'a aucun fondement théorique, qu'il soit retiré des outils qu'ils utilisent. Enfin, je vous invite à lire, ou à relire, le livre du Collectif Onze sur la justice familiale et, en particulier, sur la dimension « genrée

n'aboutisse en réalité à alourdir encore davantage la peine qui pèse sur les mères et les enfants dans tous ces cas où le juge aux affaires familiales s'est trompé. Et malheureusement ces cas-là sont nombreux ! La

donc tout d'abord un filtrage opéré par le juge aux affaires familiales, dont la mission est une mission d'équilibre et de recherche de l'intérêt de l'enfant ; il y aurait ensuite, comme vous l'avez dit, le pouvoir d'appréciation du procureur de la République, afin que

peut déjà utiliser les procédures pénales prévues en cas de non-représentation d'enfant et le faire, le cas échéant, en comparution immédiate, c'est-à-dire de manière extrêmement rapide.

Le débat se déroule hors sa présence. C'est la voie qu'il faut suivre. C'est la raison pour laquelle je soutiens la position de la commission et je vous engage à ne voter ni l'un ni l'autre de ces amendements.

Je n'ai aucun doute sur ce point et trouve que les échanges que nous venons d'avoir sont évidemment très loin d'être médiocres. Cela peut nous inciter à retravailler le texte, peut-être au cours de la navette, pour trouver la meilleure solution possible.

de demander au juge aux affaires familiales, en cas de séparation, l'attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille si les enfants y ont leur résidence habituelle, quelle

défendre notre collègue. Il vise à introduire dans le code civil des dispositions permettant aux partenaires de PACS ou aux concubins de demander au juge aux affaires familiales, en cas de séparation, l'attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille si les enfants y ont leur résidence habituelle,

à voter ces amendements. du logement de la famille dans les phases transitoires que sont les séparations peut provoquer d'importantes tensions entre les anciens concubins, dont risquent de souffrir les enfants. Pour les éviter, nous proposons d'étoffer les prérogatives du juge lorsqu'il est saisi par des couples non mariés,

Sans domicile ou lieu d'accueil, ceux-ci sont souvent exposés aux réseaux de traite des êtres humains, adoptent parfois des conduites à risque : alcool, drogue ou produits illicites. Par exemple, le cas des mineurs non accompagnés de la Goutte d'Or a particulièrement été médiatisé. Depuis l'examen du projet de loi Asile et immigration, nous réfléchissons aux moyens d'améliorer la prise en charge de ces jeunes, en lien avec la société civile. Nous souhaitions à l'origine créer la possibilité de recourir à une sorte de parrainage pour les familles françaises souhaitant accueillir ces mineurs. Les amendements que nous défendons aujourd'hui sont un peu différents, mais cherchent à atteindre le même objectif. Ainsi, l'amendement n° 302 rectifié facilite l'interprétation par le juge de la notion de désintérêt des parents en introduisant une présomption simple de désintérêt pour les parents de mineurs isolés étrangers. Cela devrait favoriser l'uniformisation des pratiques jurisprudentielles et permettre aux juges de prononcer plus facilement ces délégations d'autorité parentale au bénéfice de tiers de confiance ou de l'aide sociale à l'enfance.

ces jeunes mineurs, cette présomption nous paraît attentatoire aux droits des parents de ces enfants, quand bien même ceux-ci ne seraient pas joignables immédiatement

par le juge des enfants, voire d'organiser un transfert ponctuel de la compétence relative à la tutelle de ces mineurs au profit du juge des enfants. S'agissant ici d'une délégation d'autorité parentale et non d'une mise sous tutelle de ces enfants, il ne nous semble pas opportun de prévoir un tel transfert de compétence. Quel est l'avis

d'abandonner en délaissant leur responsabilité aux autorités. Il y a toute une question de responsabilisation des parents à régler, mais je ne pense pas que le sujet soit encore suffisamment travaillé. En tout cas, je souhaitais que l'on en prenne acte.

d'élargir le périmètre d'intervention des tribunaux de commerce pour les ériger en « tribunaux des affaires économiques ». Actuellement compétents pour les commerçants et les artisans, les tribunaux de commerce se verraient ainsi confier les procédures collectives des professions libérales, des agriculteurs et des conjoints collaborateurs. Sur le plan de l'organisation judiciaire, une telle évolution serait tout à fait importante, et c'est la raison pour laquelle elle me semble nécessiter au préalable, une étude d'impact et, d'autre part, la consultation des parties prenantes, notamment les professionnels concernés. Sur le plan juridique, l'évolution qui est proposée par la commission des lois demande à repenser la notion d'acte de commerce, voire ce qu'est le droit commercial. Enfin, celle-ci remettrait en question les spécificités du monde agricole, des professions libérales et du monde associatif.

ne correspond pas à une réalité économique. Sauf si votre intention- ce serait autre chose -est d'envisager à terme la suppression des tribunaux de commerce, ce qui représenterait une dépense nouvelle pour l'État.

une définition de la consultation juridique qui est assez proche de celle qu'en a donnée la Cour de cassation. L'actuel article 54 de la loi du 31 décembre 1971 fixe le cadre général d'exercice des activités de consultation en matière juridique et de rédaction d'actes sous seing privé, dans un objectif de protection du justiciable. Ainsi, certaines professions du droit ont la qualité pour délivrer des consultations juridiques, ce qui est le cas des membres des professions judiciaires et juridiques réglementées, notamment les avocats, les notaires ou encore les huissiers de justice. D'autres professions réglementées, par exemple les experts-comptables, peuvent également délivrer des consultations juridiques, mais uniquement dans les strictes limites qui sont autorisées par la réglementation et dans les domaines qui relèvent de leur activité principale. Pour d'autres personnes ou organismes, telles les associations, par exemple, la délivrance de consultations juridiques est au contraire subordonnée à un agrément qui permet la pratique du droit à titre accessoire, qui est accordé par un arrêté et qui fixe, le cas échéant, des conditions de qualification ou d'expérience juridique. Ce dispositif, qui est protecteur et qui est parfaitement délimité, est encore renforcé par l'article 66-2 de de la loi de 1971, qui sanctionne pénalement la pratique d'une activité juridique qui n'est pas autorisée. Il n'existe pas aujourd'hui de définition légale de la consultation juridique, mais en réalité il y a une définition stabilisée qui résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation. Il nous semble que l'introduction dans la loi, comme vous le proposez, d'une définition de la consultation juridique qui reprendrait les critères dégagés par la Cour de cassation et les précisions qu'elle a pu apporter au fil de sa jurisprudence ne modifierait pas le sens de cette jurisprudence

Par ailleurs, le dernier alinéa de l'amendement, tel que vous l'aviez rédigé, semblait réserver aux seules professions réglementées du droit l'exploitation d'un traitement numérique aux fins de délivrance d'une consultation juridique ou de rédaction d'un acte sous seing privé.

présenter l'amendement n° 23. L'article 21 étend le champ d'application du recours aux magistrats honoraires dans les juridictions administratives. Il est clair que le recours aux magistrats honoraires pour venir en appui de juridictions en sous-effectif ou qui se trouvent en tension en matière de traitement des requêtes n'est pas une mauvaise chose en soi, à condition d'en user de manière ponctuelle. Bien entendu, ce dispositif ne saurait effectivement pas remplacer le recrutement nécessaire de magistrats supplémentaires, l'apport de magistrats expérimentés poursuivant une activité juridictionnelle dans le cadre de l'honorariat ne pouvant être que subsidiaire. Il est évident que permettre aux chefs de juridiction de confier à un magistrat honoraire des fonctions d'aide à la décision apparaît comme une possibilité symboliquement désastreuse pour des magistrats par nature très expérimentés, qui se retrouveraient ainsi, dans le cadre de l'honorariat, dans une situation d'infériorité par rapport à leurs collègues en activité. Une telle possibilité ne pourrait d'ailleurs que dissuader d'éventuels volontaires. Je ne m'aventurerai pas non plus dans le détail des dispositions de cet article, mais je relève qu'une fois encore l'objectif du Gouvernement est clair à entendre les professionnels de la justice administrative, si ce genre de mesure est prise, cela n'est ni dans le but d'améliorer les conditions de travail des magistrats ni dans celui d'améliorer la qualité de traitement des requêtes d'administrés, mais bien dans le but de faire des économies sur le dos des uns et des autres. C'est pourquoi, une fois encore, nous nous opposons à cette logique purement comptable dans laquelle le service public de la justice ne saurait rester cantonné.

Cette disposition risque de produire des tensions au sein des chambres : le positionnement de ces magistrats très expérimentés comme soutien à des magistrats plus jeunes peut s'avérer délicat en pratique, ces magistrats devenant en quelque sorte des vacataires. Pourquoi ne pas rallonger quelque peu leur carrière de manière transitoire, sachant que cela ne sera plus nécessaire lorsque les recrutements suffisants auront porté leurs fruits ? Quel est l'avis de la commission ? La

à la fois pour qu'ils puissent intégrer les formations collégiales, ou bien en tant que juges uniques, ou bien pour qu'ils puissent exercer des fonctions d'aide à la décision. Ces magistrats honoraires sont extrêmement précieux, tant pour les juridictions judiciaires que pour les juridictions administratives. Je dois également préciser que ces magistrats honoraires sont très demandeurs de pouvoir intégrer ce type de fonction, et leur expérience nous est extrêmement utile. L'extension du recours aux magistrats honoraires apparaît comme une solution parmi d'autres qui permet d'accélérer le traitement des requêtes aussi bien par les tribunaux administratifs- objet de l'article 21 -que par les cours administratives d'appel. Ce recours accru aux magistrats honoraires implique bien sûr de clarifier et de renforcer les règles déontologiques et disciplinaires qui s'appliquent spécifiquement à cette catégorie de magistrats ; c'est ce que nous vous proposons de faire. Leur appui

Thani Mohamed Soilihi. Le code de justice administrative interdit la nomination au sein d'une juridiction administrative d'un conseiller qui aurait préalablement occupé certaines fonctions depuis moins de trois ans dans le ressort de celle-ci. Ce régime apparaît trop sévère et crée des contraintes excessives à la mobilité des magistrats. Un tel constat appelle à trouver un nouveau point d'équilibre entre la volonté de prévenir les conflits d'intérêts et le souhait de voir les magistrats enrichir leur connaissance de l'administration. L'amendement envisagé ne touche pas aux incompatibilités électives ; il tend juste à supprimer certaines fonctions prohibées à limiter aux collectivités territoriales de plus de 100 000 habitants celles pour lesquelles les fonctions de direction générale des services entraînent l'interdiction de nomination au sein des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Si l'amendement devait être voté et prospérer tout au long de la procédure, serait ainsi possible la nomination dans une juridiction d'un magistrat qui aurait occupé depuis moins de trois ans, dans le ressort de cette juridiction, dans le ressort de cette juridiction, la fonction de directeur régional ou départemental d'une administration publique de l'État, des fonctions de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale et des fonctions de directeur général des services d'une collectivité territoriale de moins de 100 000 habitants.

Pourquoi ? Parce que cet amendement introduit pour les conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de la souplesse

qu'il existe de manière traditionnelle dans les juridictions administratives une pratique : celle du déport. Ainsi, un magistrat administratif qui aurait à connaître d'un dossier dont il aurait dont il aurait lui-même eu à connaître auparavant dans des fonctions administratives se déporterait nécessairement. Cette pratique est couramment utilisée dans les juridictions administratives

je les comprends. Sans minimiser leur portée, j'ai presque envie de dire que ce ne serait pas la première fois que nous voterions une disposition souffrant d'une insuffisance d'évaluation.

parallélisme des formes, il apparaît opportun d'appliquer cette règle également pour les membres honoraires du Conseil d'État et les magistrats honoraires des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la Cour des comptes des chambres régionales des comptes, et de l'ordre judiciaire. Par ailleurs, à travers cet amendement, nous proposons de ratifier l'ordonnance du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant le Conseil d'État, ainsi que l'ordonnance du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

ces ordonnances avait été accordée à l'article 86 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires en même temps que l'habilitation à procéder de la même façon pour les juridictions financières. L'ordonnance relative à la Cour des comptes et aux juridictions financières a donné lieu à un véritable examen au Parlement, et le projet de loi de ratification a été définitivement adopté en août 2017.

porte diverses dispositions statutaires concernant le Conseil d'État, a consacré un droit à la formation de ses membres et a également modifié la composition et les compétences de la commission consultative, devenue la commission supérieure du Conseil d'État, afin d'en faire une véritable instance de dialogue social, mais aussi de discipline. Les garanties qui sont offertes au sein de la procédure disciplinaire applicable aux membres du Conseil d'État ont également été renforcées afin de mieux assurer leur indépendance. La seconde ordonnance, qui porte dispositions porte dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, a renforcé et approfondi l'indépendance des magistrats administratifs en modifiant la composition et les missions du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans le sens d'une plus grande indépendance et d'une plus grande autonomie de ce conseil. Cette ordonnance a encore précisé les dispositions relatives à la formation et aux affectations des magistrats administratifs, ainsi qu'à leur évaluation, et elle a créé un régime disciplinaire propre aux magistrats administratifs présentant des garanties en adéquation avec leurs fonctions juridictionnelles. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs exerce désormais directement le pouvoir disciplinaire

je vous invite à voter les deux parties de cet amendement.

Dans la même perspective que l'article précédent, l'article 22 prévoit la création du statut de juriste assistant. Le but est évident : réduire les dépenses et éviter le recrutement nécessaire de magistrats administratifs de plein exercice. Le Syndicat de la juridiction administrative explique que la multiplication des statuts de « sous-magistrat » ou de « semi-magistrat » qui auraient vocation à alléger la charge de travail des magistrats de plein exercice, et en réalité à maintenir le nombre de ceux-ci à un niveau inférieur aux besoins effectifs, n'a pour effet que de créer une justice administrative à plusieurs vitesses, avec une qualité d'expertise variable selon les contentieux et confiée à des personnes qui ne disposent pas des garanties, notamment d'indépendance, attachées à la qualité de magistrat. Encore une fois, les motifs tirés de la nécessaire maîtrise des finances publiques ne sont pas recevables en ce qui concerne l'exercice d'une mission régalienne, que cette mission précise ne concerne qu'un nombre d'agents publics relativement restreint. Nous faisons nôtre la réflexion des professionnels de la justice administrative. À nos yeux, il aurait été utile de clarifier les différents statuts de l'aide à la décision dans les juridictions administratives et de s'interroger sur l'opportunité d'une

L'article 22 reprend le dispositif prévu à l'article 24 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI siècle, relatif au recrutement des juristes assistants dans les juridictions de l'ordre judiciaire. Certes, dans le cadre de l'examen de cette loi, la commission s'était opposée à la création d'un statut supplémentaire de personnels. À son sens, cette création risquait de rendre peu lisible la répartition des compétences entre les différents intervenants. Néanmoins, ce nouveau statut a tout de même été créé, et les magistrats judiciaires semblent pleinement satisfaits du concours des juristes assistants. Dès lors, il n'y a pas de raison, nous semble-t-il, de s'opposer à leur déploiement au sein des juridictions administratives. J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement. Madame la sénatrice, l'avis du Gouvernement

De ce point de vue, la possibilité ouverte par le présent texte de recruter à temps partiel des personnes titulaires d'un master 2 en droit et dotées de deux ans d'expérience ne nous paraît pas acceptable. Lors de nos auditions, il nous a été dit que le salaire proposé pour un poste de juriste assistant est de 1 800 euros, ce qui n'apparaît pas excessif au regard des qualifications requises et des responsabilités endossées. Si ces personnes étaient recrutées à mi-temps, elles percevraient un salaire de 900 euros, ce qui les placerait sous le seuil de pauvreté défini en France. Cette éventualité n'est pas acceptable. Au-delà du risque d'enfermer ces personnes qualifiées dans des fonctions sous-rémunérées,

cet amendement était adopté, l'on supprimerait la possibilité de nommer des juristes assistants à temps incomplet dans les juridictions administratives.

doit s'inscrire dans une stratégie de long terme pour ces juridictions comme pour les personnes ainsi recrutées. Nous considérons donc que des voies particulières de recrutement interne doivent être réservées Les juridictions ont tout à y gagner. Il s'agit d'un moyen indéniable de recruter des personnes déjà formées à la rédaction de décisions, connaissant le fonctionnement d'un tribunal et de l'administration en général. De plus, ce

ne sont pas forcément très bien représentés à l'ENA. La nature de la fonction de juriste assistant justifie, à nos yeux, de pouvoir réduire de quatre à trois ans la durée d'exercice requise, du fait des qualifications particulières acquises par ces personnes.

d'exercice. On ne précise pas le type de fonctions que les juristes assistants auraient dû occuper pendant ces trois années. De plus, il n'y a pas de raison de prévoir une durée d'exercice de leurs fonctions inférieure à celle qui est exigée pour les agents publics,

avec trois ans d'ancienneté seulement.

La bonne administration de la justice ne suppose-t-elle pas de répartir équitablement les moyens entre les justiciables ? Quel est l'avis de la

à une formation de trois juges des référés pour traiter des contentieux administratifs de référés en matière précontractuelle et contractuelle, qui se caractérisent par leur complexité et leurs forts enjeux économiques, est évidemment un gage d'amélioration de la qualité et de l'efficacité de la justice

à établir une distinction parmi les membres de la commission du contentieux du stationnement payant, entre, d'une part, les membres permanents et, d'autre part, les membres non permanents. Enfin, cet amendement vise à ratifier deux ordonnances de 2015 liées au contentieux du stationnement payant. Là aussi, le travail de dépoussiérage doit être continué. Quel est l'avis de la commission ? Au travers

lorsqu'il a examiné la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, ou loi SILT. Cette censure partielle concerne la procédure de renouvellement des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, Ces dispositions prévoyaient que le renouvellement des mesures de surveillance devait intervenir cinq jours avant leur entrée en vigueur, afin que les intéressés puissent saisir dans les quarante-huit heures le juge des référés du tribunal administratif, à charge pour celui-ci de statuer dans les soixante-douze heures. Or le Conseil constitutionnel a considéré que l'office du juge des référés, limité au contrôle des atteintes graves et manifestement illégales à une liberté fondamentale, était insuffisant, et que ce contrôle devait, au contraire, porter sur la régularité et le bien-fondé de la décision de renouvellement. Il est donc proposé de s'inspirer de la procédure contentieuse applicable aux mesures d'éloignement notifiées aux personnes placées en rétention administrative.

heures. Le Conseil constitutionnel a également censuré les délais de deux mois et de quatre mois qui étaient laissés au juge administratif pour statuer sur la légalité des mesures individuelles initiales. En conséquence, nous proposons de diviser par deux les délais de jugement initialement prévus, en les fixant respectivement à un mois, dans le cadre de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, et à deux mois, dans le cadre de l'article L. 228-5 du même code. Dans les deux cas, le délai de saisine du juge est fixé à un mois. Enfin, le présent amendement vise à introduire un nouvel article au sein du code de justice administrative, afin de prévoir la détermination des modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance et de prévoir un décret en Conseil d'État pour leur application.

des conclusions du rapporteur public. En l'occurrence, il s'inspire d'une procédure applicable aux mesures d'éloignement qui sont notifiées aux personnes placées en rétention administrative, figurant dans le code

dont sont saisis les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. Elle ne justifie pas que, pour toutes les affaires qui leur sont soumises, un rapporteur public développe, à l'audience, ses conclusions orales.

C'est pourquoi, dans le respect des droits de la défense, le rapporteur public doit démontrer publiquement que les mesures de contrainte sont justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public. En conséquence, En conséquence, nous proposons de supprimer la mention selon laquelle l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. Nous préconisons également d'harmoniser les délais de jugement à un mois pour le régime complet et les obligations complémentaires, afin de respecter fidèlement la jurisprudence constitutionnelle, en vertu de laquelle « le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge administratif soit tenu de statuer sur la demande d'annulation de la mesure dans de brefs délais ».

amendement maintient un délai de saisine de la juridiction administrative limité à un mois, alors même que cette limitation a été expressément censurée par le Conseil constitutionnel. Il serait sans doute plus raisonnable d'envisager des délais de saisine de deux mois, jours fixés à la juridiction pour statuer. Ensuite, contrairement aux dispositions du CESEDA dont il s'inspire, cet amendement ne prévoit pas la présence de l'intéressé à l'audience. Notre sous-amendement vise à réparer ces omissions. En outre, il prévoit

le territoire français, ou OQTF, lorsque l'étranger est placé en rétention. Comme pour ce type de recours, les décisions de renouvellement des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance présentent un caractère d'urgence,

j'ajoute que les moyens soulevés peuvent l'être jusqu'à l'audience. Quant à la seconde modification proposée, elle ne me semble pas davantage adaptée type de recours dont il est ici question. L'amendement du Gouvernement tend à diviser par deux les délais de jugement initialement prévus, en les fixant respectivement à un et deux mois, contre deux et quatre mois. Il n'apparaît pas souhaitable d'harmoniser les délais de jugement à un mois. Non seulement les deux types de décisions dont

il s'agit d'imposer la présence du requérant à l'audience, excepté lorsqu'un sauf-conduit ne peut être délivré par le ministère de l'intérieur, ou, dans cette hypothèse, une représentation obligatoire par avocat. Il me semble que cette modification relève du domaine réglementaire. En tout état de cause, les dispositions actuelles du code de la sécurité intérieure dont nous discutons ne font pas, en droit, obstacle à la présence du requérant, comme c'est le cas pour n'importe quel recours pour excès de pouvoir.

de la censure partielle prononcée par le Conseil constitutionnel en mars 2018. Le Conseil constitutionnel a partiellement censuré la possibilité de procéder à la saisie des objets et documents

sur celui qui est issu de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, la saisie des autres documents et objets n'obéissait à aucune formalité particulière.

aux exigences formulées par le Conseil constitutionnel. La saisie de documents autres que des données informatiques peut en effet s'avérer nécessaire, notamment en cas de documents rédigés en langue étrangère ou de documents volumineux, en raison de l'impossibilité de les exploiter sur place. En revanche, le rétablissement des dispositions relatives à la saisie des objets apparaît inutile : d'une part, leur saisie en police administrative n'est pas nécessaire, présence relatée dans les procès-verbaux suffisant à établir les raisons sérieuses exigées par la loi ; d'autre part, lorsque leur possession est de nature à caractériser un délit, leur saisie se déroule en procédure incidente, selon les règles de la procédure pénale.

dix ans. Cette avancée sera vraisemblablement utile aux victimes ne pouvant se déplacer ou redoutant de se déplacer pour porter plainte. Le dépôt de plainte représente une charge administrative importante pour les forces de l'ordre dans les commissariats et les gendarmeries, mais également une épreuve pour certaines victimes. Pour autant, la faculté de porter plainte en gendarmerie ou au commissariat doit être maintenue pour les victimes ayant fait la démarche de s'y rendre. Tel est l'objet de cet amendement.

Ce titre comporte des mesures très disparates et d'intérêt inégal, sur lesquelles nous reviendrons, mais il marque une volonté générale : l'accroissement des pouvoirs du parquet, une marginalisation de l'information judiciaire, une simplification et une réduction des garanties et une forme de défiance vis-à-vis du juge, avec un statut du parquet dont nous savons qu'il n'est toujours pas modifié et qui fait évoluer de manière implicite notre système vers, peut-être, un système anglo-saxon. Nous sommes préoccupés par cette simplification, qui a vocation à accroître les pouvoirs du parquet sans contrôle, à faciliter le recours à des techniques spéciales et à banaliser des procédures normalement réservées à l'état d'exception. Nous sommes inquiets

Vous souhaitez multiplier par deux la durée de l'enquête de flagrance, à laquelle correspondent des pouvoirs exorbitants permettant des géolocalisations ou des interceptions judiciaires. Vous souhaitez également étendre les possibilités de perquisition à un plus grand nombre de délits,

De même, s'il s'agit de faits graves ou exigeant une audition de la victime, la plainte en ligne sera nécessairement suivie de l'audition de la victime par les enquêteurs. La plainte en ligne constitue ainsi une première démarche,

n° 291 rectifié. Compte tenu de la volonté de développer la dématérialisation des plaintes, il est important de préciser explicitement l'interdiction pour les forces de l'ordre en charge du recueil des plaintes dans les services de police nationale et les unités de gendarmerie nationale de refuser le dépôt sur place, au motif que la victime pourrait porter plainte en ligne. Il s'agit seulement de simplifier le parcours judiciaire des victimes et de protéger les personnes dépourvues de connaissances numériques, tout en permettant le développement d'outils de nature à faciliter le travail des forces de l'ordre.

Peut-être pourrons-nous, dans le cours de la navette, affiner notre rédaction- nous n'y sommes pas opposés. Mais je ne pense pas que cela soit une excellente idée de permettre d'emblée une plainte en ligne pour l'ensemble des infractions.

« Il paraît excessif de prévoir que n'importe quelle infraction, y compris par exemple un crime ou un délit grave contre la personne, puisse faire l'objet d'une plainte en ligne

Il nous avait semblé, à la lecture de l'étude d'impact, que la plainte en ligne viserait d'abord des escroqueries sur internet ou des fraudes à la carte bancaire, sans préjudice d'un futur élargissement de cette nouvelle procédure, si elle fait la preuve de son efficacité.

La plainte en ligne est réellement, pour nous, un outil facilitateur pour les victimes. Elle leur permet soit rapidement un contact, soit d'éviter d'avoir à se déplacer et, dans des cas très précis- je pense notamment aux violences

la possibilité- ce n'est qu'une possibilité -de déposer plainte en ligne. Il nous semble extrêmement important de prévoir cette autre voie d'accès au juge. Une plainte en ligne sera évidemment suivie d'un contact physique avec un agent qui,

Je ne sais pas s'il y a des pratiques divergentes, mais il y a un texte qui garantit le droit des victimes à être entendues par les commissariats où elles se présentent. Il s'agit,

au contraire, être mis en responsabilité dès le début de la procédure. C'est pourquoi nous proposons la mention des poursuites encourues en cas d'usage dévoyé de cet outil préalablement au dépôt de la plainte. Une utilisation dévoyée de la plainte en ligne rendrait aussi plus difficile la tâche des forces de l'ordre en charge de trier et de traiter ces plaintes.

que l'institution de la plainte en ligne dans certains contentieux ne devienne le prétexte à des pratiques plus ou moins institutionnalisées de refus illicite de prise de plaintes de la part de services de police et de gendarmerie qui seraient désireux de soigner leurs statistiques, en renvoyant les victimes sur des plateformes en ligne à l'accessibilité et à l'efficacité aujourd'hui totalement virtuelles.

être déposée selon les règles générales du code de procédure pénale. Cette précaution passe par l'insertion à l'article 15-3-1 de ce code d'un d'un alinéa garantissant expressément que le recours à la plainte en ligne ne peut pas être imposé à la victime. De plus, dès lors qu'un décret devra préciser dans quels cas la plainte en ligne sera autorisée, il paraît utile de fixer ce principe dans la loi. Quel

et il est contraint d'ordonner le renvoi si cette formalité n'a pas été accomplie. En imposant au tribunal correctionnel de renvoyer l'affaire à une audience sur les intérêts civils lorsqu'il a statué sur l'action publique, sans qu'il soit établi que la victime ait été avisée de la date d'audience, le présent projet de loi altère le statut des victimes. Selon nous, il s'agit d'une atteinte aux droits En effet, comment peut-on envisager, au vu des impératifs du droit à un procès équitable, de permettre à un jugement correctionnel d'intervenir à l'insu de la victime ? De plus, la condition prévue par le projet de loi autorisant le tribunal a passé outre l'avis à victime lorsqu'il estime que la présence de celle-ci n'est pas indispensable au débat repose sur un critère d'appréciation très large, laissé au seul arbitrage du tribunal, ce qui pose problème, d'autant que la question est insusceptible de recours de la part de la victime évincée. Les répercussions négatives que cette mesure risque d'entraîner n'ont sans doute pas été suffisamment prises en considération, qu'il s'agisse du fonctionnement des services du greffe et des formations chargées des intérêts civils. Les avis à victime constituent une charge nécessaire, mais lourde pour les services du greffe, de la police et de la gendarmerie, qui sont, par ailleurs, soumis à d'importantes contraintes en termes de moyens. Il est donc à craindre que, dans certains services, cette disposition n'entraîne un désinvestissement de fait sur ce champ, conduisant l'absence d'avis à victime, aujourd'hui signe d'un oubli ou d'un dysfonctionnement ponctuel, à devenir une pratique généralisée aux dépens des victimes. Enfin, la pratique du renvoi systématique devant les formations chargées des intérêts civils est de nature à engorger celles-ci dans des proportions au moins équivalentes au temps gagné devant le tribunal correctionnel.

d'inciter les tribunaux à priver la victime de sa participation au procès, en renvoyant le jugement de l'action civile, alors même que la victime n'aurait pas été convoquée. La loi impose d'aviser la victime de l'audience et, si cela n'a pas été fait, le dossier doit être renvoyé. Nous ne changeons pas cette règle. C'est uniquement dans les cas où l'avis à victime a bien été adressé à cette dernière- en pratique par lettre simple mais que celle-ci n'est pas présente et qu'il n'est pas certain qu'elle ait eu connaissance de cet avis que le renvoi de l'affaire sur l'action civile est prévu. Cela évitera ainsi, selon nous, à la victime de découvrir après l'audience qu'une condamnation pénale a été prononcée en son absence et qu'elle doit elle-même intenter un procès civil devant le juge civil pour être indemnisée. Madame la sénatrice, monsieur le rapporteur Buffet, si la rédaction que je propose est ambiguë, si vous estimez qu'elle peut être précisée, je veux bien la retravailler. Peut-être également faut-il transformer l'obligation de renvoi prévue par le texte en une simple possibilité, afin d'assouplir le dispositif Je suis prête à revoir ce texte à l'Assemblée nationale pour qu'il soit amélioré sur ces points, mais l'amendement de suppression proposé me semble devoir être rejeté. Je le dis fondamentalement, cette mesure est favorable aux victimes,

est à Mme Laurence Harribey. Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 13 de l'article 26. L'ajout de la possibilité pour la victime de se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel par voie de communication électronique constitue clairement un ajout bienvenu, dans la mesure où ce mode de saisine est prévu comme une possibilité supplémentaire. Néanmoins, les dispositions envisagées pour l'alinéa 2 de l'article 420-1 du code de procédure pénale présentent une difficulté au regard du respect des droits de la défense. En effet, s'il peut paraître tentant de supprimer un délai de recevabilité pouvant être perçu comme rigoureux, il convient de relever qu'un délai est rendu impératif par la nécessité de mettre la défense en mesure de répondre à la constitution de partie civile. Or la rédaction envisagée pour l'alinéa 2 de cet article conduirait à permettre au tribunal correctionnel de statuer sur une constitution de partie civile dont la défense n'aurait pas eu préalablement connaissance, et ce en violation de la notion de droit à un procès équitable.

au moyen d'une communication électronique et que cette constitution de partie civile est recevable dès lors qu'elle aura été reçue avant les réquisitions du ministère public. Cela constitue une avancée.

un avis défavorable, madame la sénatrice, pour les raisons précises que vient d'énoncer M. le rapporteur. Cette partie du texte est évidemment très favorable aux victimes.

Le sujet est techniquement délicat. Je peux comprendre- et notre rapporteur a raison de le dire -que le tribunal reçoive par voie électronique, peut-être même au début de l'audience, la constitution de partie civile. Il faut permettre au prévenu et à son avocat d'en prendre connaissance et de pouvoir y répondre,

Aujourd'hui, ce droit n'existe pas : la victime peut certes faire appel sur ses intérêts civils, mais elle ne peut pas demander la tenue d'un second procès pénal, qui pourrait aboutir à l'établissement de la culpabilité pénale du mis en cause. est souvent vécue comme un second traumatisme pour la victime. Car une décision d'acquittement ne signifie pas seulement que son agresseur présumé est innocenté : aux yeux de la société, c'est la victime elle-même qui devient une menteuse potentielle, ce qui est particulièrement ravageur dans les cas de violences sexuelles, parfois difficiles à prouver matériellement. Il faut s'imaginer la détresse d'une victime qui voit le ministère public requérir une très lourde peine, puis ne pas faire appel de l'acquittement prononcé par la cour. Et cet exemple n'est pas isolé : entre 2003 et 2005, les cours d'assises d'appel n'ont eu à juger que 76 affaires dans lesquelles un acquittement avait été prononcé, alors que le nombre d'acquittements annuel dépasse les 200- il était de 250 en 2006. Il ne fait donc pas de doute que la majorité des acquittements n'est pas frappée d'appel par le parquet. Le droit d'appel de la victime en cas de relaxe serait en outre le prolongement naturel et cohérent des droits dont bénéficient actuellement les victimes. En effet, la victime déclenche l'enquête en portant plainte, peut passer outre un classement sans suite du procureur par une constitution de partie civile et a la capacité de faire appel des ordonnances de non-lieu du juge d'instruction. C'est pourquoi des magistrats éminents, comme Claude Mathon, avocat général près la Cour de cassation, ont pu défendre l'idée que le droit d'appel de la victime en cas de relaxe ou d'acquittement constituerait une mise en cohérence de notre système juridique. Quel est l'avis de la commission

de notre justice pénale, pour une raison simple : celui qui exerce les poursuites et demande la sanction, c'est le procureur de la République ou l'avocat général, donc le ministère public. Au nom de l'État, il demande la sanction et requiert à l'audience. La victime est bien sûr présente à l'audience, mais elle est là pour obtenir réparation civile du dommage

Le magistrat, le juge décide évidemment et les possibilités d'appel ne sont alors ouvertes qu'au procureur de la République ou au condamné lui-même, la victime ne pouvant pas elle-même faire appel, ce qui pourrait s'apparenter à certains égards à une forme de justice privée.

que la cour d'assises ou le tribunal correctionnel apparaissent à un moment ou à un autre comme un lieu où la vengeance privée s'exprime. Il est vraiment important de laisser la possibilité d'interjeter appel au ministère public.

est évidemment défavorable. Aller dans le sens proposé constituerait une véritable révolution juridique, qui n'est en aucun cas conforme à notre droit. L'article 1 du code de procédure pénale donne à la victime le droit de mettre en mouvement l'action publique, ce qui est logique où ce droit est la contrepartie du pouvoir de classement en opportunité du ministère public. Mais notre droit n'a jamais permis à la victime d'exercer elle-même l'action publique, ce rôle étant évidemment confié aux seuls magistrats du parquet, comme vient de le dire M. le rapporteur. J'ajoute que, en pratique, le fait de permettre aux victimes de faire appel des acquittements prononcés par les cours d'assises, alors même que le parquet aurait estimé ne pas pouvoir faire appel, ne répondrait évidemment pas aux objectifs. Comment peut-on imaginer un instant, alors que le le ministère public lui-même estimerait l'appel inutile, que les cours d'assises pourraient déclarer l'accusé coupable ? D'ailleurs, en matière d'assises, il est prévu que seul le procureur général puisse faire appel d'un acquittement, ce pouvoir n'étant même pas donné au procureur de la République. Comme vous le voyez, madame la sénatrice, l'appel doit être interjeté avec beaucoup de discernement. On ne peut donc pas donner un tel pouvoir à la victime elle-même. Les conclusions sont identiques pour l'amendement suivant en matière correctionnelle.

pénale organisent selon certaines modalités la protection des témoins, rien n'existe actuellement- je dis bien : rien -pour les victimes d'infractions qui ne souhaitent pas révéler leur propre identité. C'est notamment le cas pour certaines catégories d'agents publics particulièrement exposées aux agressions : le fait de devoir décliner son identité est peu incitatif pour déposer plainte. L'objet de cet amendement est d'ouvrir la possibilité à l'administration de faire écran entre l'auteur des faits et son agent, permettant ainsi que l'identité de l'agent n'apparaisse pas en tant que telle. Ainsi, Ainsi, les agents publics pourront déposer plainte de façon anonyme lorsqu'ils sont victimes d'agressions. de la commission ? Cet amendement prévoit d'autoriser les personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public à déposer plainte anonymement, dans le but de les protéger d'éventuelles représailles. Le problème soulevé à travers cet amendement est réel ; il n'y a aucun doute sur ce point : des policiers ou des gendarmes notamment, mais aussi des enseignants ou des agents hospitaliers, pour ne citer que ces quelques exemples, peuvent être victimes d'agressions dans le cadre de leurs fonctions, et les craintes de représailles sont réelles. Cependant, l'anonymat cadre mal avec certaines exigences de la procédure pénale : comment organiser éventuellement une la victime et l'auteur des faits sans dévoiler l'identité de celle-ci ? Par ailleurs, il est à craindre que la protection apportée par l'anonymat ne soit, dans bien des cas, relative. On peut imaginer de nombreux cas où il sera très facile, pour ne pas dire extrêmement simple, de pouvoir déterminer

le dispositif prévu en matière pénale comporte un certain nombre d'instruments : l'interdiction de paraître dans certains lieux ou d'entrer en relation avec certaines personnes, voire le placement en détention provisoire pour les personnes les plus dangereuses. C'est la raison pour laquelle la commission des lois souhaiterait, madame

et pour partie satisfait. Excessif, parce que, d'une manière générale, la qualité de victime permet difficilement de conserver un anonymat dans la procédure, dès lors qu'il s'agit d'une partie qui demande l'exercice d'un droit. Pour partie satisfait, parce que l'objectif que vous poursuivez au travers de votre amendement trouve déjà des réponses dans le droit positif. Je pense notamment, madame la sénatrice, à l'article 15-4 du code de procédure pénale qui permet déjà aux enquêteurs- policiers, gendarmes et, par assimilation, douaniers -d'être identifiés dans les procès-verbaux d'enquête par un numéro lorsqu'il existe des risques d'atteinte à leur vie privée ou à leur intégrité ou à celle de leurs proches. Cet article permet également à ces enquêteurs, lorsqu'ils ont été autorisés à s'identifier par un numéro, de conserver ce mode d'identification s'ils se constituent parties civiles en raison d'une infraction dont ils auraient été victimes dans l'exercice de leur mission. C'est la raison pour laquelle je vous propose également, madame la sénatrice, de retirer votre amendement, sinon je me verrai dans l'obligation d'émettre un avis défavorable.

tel qu'il en existe déjà à l'étranger. Depuis vingt-cinq ans, on développe ce système aux États-Unis, ce qui permet d'y suivre 90 % de la population carcérale. Ce système offrirait en effet une meilleure information et protection des victimes, une simplification des textes, un allégement des coûts. Cette solution permet à une victime de connaître le statut carcéral de son agresseur pratiquement en temps réel : s'il est incarcéré, s'il est transféré, tout ce qui touche l'application de la sentence. pleinement dans la démarche de modernisation, de simplification et de rationalisation des coûts voulue par le Gouvernement dans le cadre de cette loi de programmation pour la justice. Elle permettrait enfin de pallier une situation génératrice d'angoisse pour les victimes, une situation dénoncée encore récemment par une partie de la doctrine juridique- Léa Castellon, partie de la doctrine juridique- Léa Castellon, « [ ...] Lorsque les mesures d'aménagement de peine ne sont pas assorties d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile ne bénéficie que d'un éventuel droit à l'information. [ ...] La décision d'informer la victime est laissée à la libre appréciation des juridictions d'application des peines, la victime ne peut donc pas se plaindre d'un manque d'information. Or, au regard de la sécurité de certaines victimes et du risque de récidive, il est nécessaire que la victime obtienne automatiquement, dès qu'elle en émet le souhait, des informations sur les conditions de sortie du condamné.

qui vise seulement la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté. Les permissions de sortir seront désormais concernées. Cette amélioration de l'information des victimes nous a paru être une préoccupation légitime. Quel est l'avis du Gouvernement ?

du code de procédure pénale, qui prévoit déjà, dans certains cas, l'information de la victime en cas de libération d'un condamné. En effet, cet article dispose que, si le condamné se trouve en présence de la victime et si, au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l'intéressé, il apparaît qu'une telle rencontre doit être évitée, les juridictions de l'application des peines doivent assortir les décisions de libération d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, d'une interdiction de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail. Le prononcé de cette interdiction est d'ailleurs obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour des infractions de nature sexuelle ou pour des violences graves, qui sont visées par le code de procédure pénale. La victime est donc avisée de la libération et de cette interdiction de contact, sauf si elle a fait connaître qu'elle ne le souhaitait pas. Parce que des dispositions sont déjà prévues et me semblent suffisantes, je ne suis pas favorable à l'amendement que vous proposez,

ainsi libellé : La parole est à M. Henri Leroy. Cet amendement vise à donner une place plus importante aux victimes au stade de l'application de la peine. Parce que la protection physique de la victime est parfois en jeu et que sa reconstruction psychologique passe par l'exécution complète de la peine, il importe que celle-ci puisse être présente, ou représentée, lors de toute décision tendant à libérer le condamné avant la fin de sa peine. Il est utile de faire participer la partie civile aux débats contradictoires précédant les jugements de première instance des juridictions d'application des peines relatifs aux mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et de suspension de peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle, mais également aux décisions de relèvement de la période de sûreté. Ce dispositif permettrait par ailleurs de revenir sur la suppression, en 2009, des dispositions issues de la loi Clément du 12 décembre 2005 desquelles l'avocat de la victime peut faire valoir son point de vue sur les décisions d'allégement et d'aménagement de peine relevant du tribunal de l'application des peines. Le dispositif proposé est toutefois plus large que les dispositions précitées, car il porte sur toutes les mesures d'aménagement de peine, qu'elles relèvent du juge de l'application des peines, en référence à l'article 712-6 du code de procédure pénale, ou du tribunal de l'application des peines, en vertu de l'article 712-7 du même code. En outre, l'article 712-13 est modifié afin que l'avocat de la partie civile puisse aussi faire valoir ses observations lors du débat contradictoire dans le cadre de l'appel des décisions des juridictions de l'application des peines. Si la victime ne peut faire appel des décisions des juridictions de l'application des peines, elle se voit toutefois accorder le droit d'y faire valoir ses observations par le biais de son avocat, à l'instar du condamné. Enfin, dans un souci de coordination, le dernier alinéa de l'article 730, devenu inutile et redondant, est supprimé.

générale, nos concitoyens, aient parfaitement confiance dans notre dispositif judiciaire, il faut que les peines prononcées par les tribunaux puissent être exécutées rapidement et dans les meilleures conditions possibles. Nous pensons que c'est là la ligne de force qu'il faut suivre. C'est la raison pour laquelle, sur ces deux amendements, la commission

garde des sceaux. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, c'est un amendement important que je vous présente. Il vise à accélérer l'indemnisation des victimes d'attentats terroristes. Ces victimes, qui ont évidemment vécu des situations dramatiques, très douloureuses, sont aujourd'hui confrontées à un parcours procédural extrêmement complexe lorsqu'elles sollicitent la réparation des préjudices subis, ce parcours s'inscrivant aujourd'hui dans le sillage de la procédure pénale. En effet, de multiples acteurs sont susceptibles d'intervenir pour assurer cette indemnisation en fonction de l'état de la victime et également de l'avancement des investigations. Interviennent ainsi le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme, le juge d'instruction, le juge civil statuant en référé ou au fond, la juridiction pénale de jugement. Je souhaite que cette complexité procédurale ne vienne pas s'ajouter à l'épreuve qu'ont déjà subie ces victimes. C'est pourquoi j'ai demandé à Mme Chantal Bussière d'évaluer les dispositifs existants et d'identifier les améliorations susceptibles d'être apportées au parcours procédural des victimes. Mme Bussière, magistrate, m'a rendu ses conclusions il y a quelque temps, et ce sont ces conclusions, qu'elle a pu établir à la suite d'un très large processus de dialogue et de consultation, qui conduisent le Gouvernement à vous proposer l'amendement dont il est ici question. Prenant, donc, appui sur ces travaux, je vous propose de simplifier le parcours des victimes d'actes de terrorisme, d'accélérer leur indemnisation et de favoriser l'égalité de traitement entre elles. Tels sont les trois objectifs que je poursuis : simplification, accélération de l'indemnisation et égalité dans le traitement. Il ne s'agit évidemment pas ici de remettre en cause le dispositif amiable de l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, qui est assuré par le FGTI, le fonds de de renforcer son efficacité, d'y adosser un recours juridictionnel unifié et spécialisé et de veiller à une meilleure articulation avec la procédure judiciaire. Ainsi, outre le choix du médecin sur une liste d'experts, qui est prévu par le présent amendement, je vous indique dès à présent que les mesures réglementaires viendront renforcer les garanties offertes aux victimes pendant le déroulement de l'examen médical qui est pratiqué de manière systématique à la demande du FGTI, pour les rapprocher de celles qui sont offertes par la procédure civile- je pense notamment à la remise d'un prérapport ou au renforcement du contradictoire. S'agissant donc du présent amendement, afin de favoriser un traitement plus rapide et plus juste sur l'ensemble du territoire, un juge civil sera spécialisé au tribunal

Il s'agit au contraire de donner aux victimes un accès à un juge civil spécialisé, suivant en cela les recommandations qui ont été formulées par le Défenseur des droits. L'accès à ce juge se fera selon une procédure adaptée à la complexité des demandes liées à la réparation de ces préjudices très particuliers, et le traitement de ces demandes, ainsi conçu, ne retardera plus le déroulement de l'information judiciaire et la tenue du procès, qui constituent très souvent une étape indispensable dans le parcours de reconstruction de ces victimes. Cette compétence exclusive donnée au JIVAT aura pour corollaire l'incompétence des juridictions pénales pour connaître de l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction résultant d'un acte de terrorisme. Mais je tiens à souligner avec force que cette incompétence matérielle ne retirera aucun droit aux victimes d'actes de terrorisme celles-ci conserveront bien entendu toute leur place dans le procès pénal, se constituant partie civile afin soit de mettre en mouvement, soit de soutenir l'action publique. Les victimes continueront ainsi d'avoir accès au dossier de la procédure et, bien entendu, elles pourront formuler toute demande d'acte utile à la manifestation de la vérité afin de soutenir l'action publique. Il est évidemment impensable- et il n'est en aucun cas envisagé -que la parole publique ne puisse pas être portée devant le juge pénal, tant par leur témoignage direct que par la voix de leur avocat. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, cet amendement, avec la création du JIVAT, a en réalité pour objet d'accélérer l'indemnisation des victimes, cette rapidité étant évidemment liée au fait que l'indemnisation sera décorrélée du procès pénal, qui est souvent extrêmement long.

Le droit applicable aujourd'hui prévoit que les victimes de tels actes disposent d'un délai de dix ans pour demander une indemnisation de leurs préjudices corporels auprès du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, le FGTI, dans le cadre d'une indemnisation au caractère amiable, prise en charge au titre de la solidarité nationale. Sans créer de nouvelle juridiction, l'amendement tend, en premier lieu, à attribuer compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris pour connaître des demandes formées en matière de réparation du dommage corporel subi par les victimes d'actes de terrorisme. Seraient concernés

contestation du montant de l'indemnisation, contestation de l'examen médical- seraient y compris concernés, d'ailleurs, des recours subrogatoires en remboursement des indemnités ou provisions versées à la victime.

; en cas de désaccord de la victime avec ce qui est proposé, deux voies de recours s'offrent à elle : soit devant le TGI de Créteil, qui correspond au tribunal compétent du lieu du siège du fonds, soit devant le tribunal de grande instance du lieu de l'attentat. De surcroît, cet amendement vise à mettre fin aux compétences concurrentes du juge civil et du juge pénal pour apprécier l'indemnisation du préjudice résultant d'une infraction constituant un acte de terrorisme. Le juge pénal ne pourrait donc plus être saisi d'une demande en réparation d'un préjudice résultant d'une infraction de cette nature, puisque seul le nouveau JIVAT serait compétent pour examiner les demandes. Ce dispositif, par ses objectifs, nous paraît intéressant

Or- il faut dire les choses telles qu'elles sont -il existe déjà un point d'entrée unique pour l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, puisqu'il s'agit d'une procédure amiable traitée par le FGTI,

dans le ressort duquel est situé le lieu de l'attentat. Par ailleurs, le parquet de Paris disposant d'une compétence concurrente en matière de terrorisme, il est fort probable que le procès de l'auteur de l'infraction se déroule à Paris. Que l'indemnisation en matière civile soit aussi traitée par un juge affecté au TGI de Paris aurait alors, dans ces conditions, toute sa cohérence. De plus, le tribunal de grande instance de Paris dispose déjà- il faut le signaler -d'un pôle spécialisé dans la réparation des préjudices corporels, contentieux particulièrement technique auquel serait rattaché le nouveau JIVAT. La procédure d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme consiste essentiellement- il faut le rappeler, c'est important -dans des expertises destinées à évaluer les préjudices. La centralisation de la juridiction ne serait donc pas en elle-même un problème, dès lors que les victimes auraient accès à un expert

L'incompétence des juridictions pénales pour statuer sur les demandes indemnitaires nous semble également opportune. En effet, actuellement, les juridictions pénales sont compétentes pour connaître de l'action en réparation des dommages causés par une infraction qui constitue un acte de terrorisme. Or, en raison des nombreuses victimes d'un même acte terroriste, des informations judiciaires est retardé. Selon les éléments dont nous avons pu avoir connaissance, la déconnexion entre les actions pénale et civile devrait permettre de désengorger les cabinets d'instruction

entre les victimes. Ce qui nous importe, au total, c'est que le dispositif soit efficace, au service d'une réparation équitable et juste pour les victimes d'infractions terroristes. En revanche, madame la ministre, nous serons attentifs à ce que le Gouvernement mette en oeuvre les moyens nécessaires afin de faciliter autant que possible l'accès à ce nouveau juge civil tout en organisant les fameuses expertises d'évaluation des préjudices corporels au plus près de ceux et celles qui ont souffert de tels attentats. Pour toutes ces raisons- je le redis -, la commission des lois a, ce matin, émis un avis favorable

il faut d'abord imposer au fonds des délais et des obligations, comme il en existe en matière d'assurance depuis la loi Badinter de 1985- dans un temps donné, la compagnie d'assurance doit faire à la victime une offre au moins provisionnelle.

chaque situation de victime est très particulière. L'indemnisation du préjudice moral peut être uniformisée ; mais l'indemnisation du préjudice matériel, du préjudice professionnel, des pertes de chance, etc. doit être très individualisée- de telles procédures, d'ailleurs,

d'affaires. Aujourd'hui, on constate que les délais sont très longs, et que les procédures d'indemnisation n'en finissent pas. Pour les victimes, c'est intolérable. La justice est lente

de la Gontrie, pour explication de vote. Vous l'avez compris, madame la ministre : nous avons réfléchi, écouté- nous avons eu peu de jours pour cela -, et nous vous avons entendue. M. le rapporteur a parfaitement résumé les réflexions que nous avons échangées au sein de la commission des lois.

d'abord m'expliquer, d'un demi-mot, sur la procédure : il est vrai que cet amendement vous a été transmis tardivement. Vous savez, si vous avez un peu suivi l'élaboration du projet de loi que je vous présente,

À l'une des questions qui ont été posées, je répondrai que le FGTI continuera, bien sûr, de faire des offres de provision

[ ...]. Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices.

avec la création à la fois d'un juge de l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'un parquet national antiterroriste. Cette spécialisation de toute la chaîne est évidemment importante : elle ira de l'instruction au jugement, et jusqu'à l'exécution des peines. L'idée est de créer une communauté de magistrats professionnels qui soient spécialisés en matière de terrorisme, au civil comme au pénal, et qui puissent prendre en charge cette dimension si particulière de notre action judiciaire.

ont même pu obtenir des avancées -, sur la justice pénale, il semblerait que tout se soit déroulé ailleurs qu'à la Chancellerie. Cela a notamment fait dire à Basile Ader, vice-bâtonnier de Paris, que ce projet de loi était un texte « Collomb-Molins Cet article 27, premier d'une longue série, en est bien l'illustration. Il vise à étendre le recours à la géolocalisation et aux interceptions par voie de communication électronique, comme c'est déjà le cas en matière de criminalité et de délinquance organisée, lors d'enquêtes préliminaires et de flagrance sur les crimes et délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement. Alors que l'économie générale du dispositif devait conduire le législateur à s'interroger sur son maintien ou, à tout le moins, à contrôler plus strictement son utilisation, le projet de loi entend à l'inverse banaliser les interceptions téléphoniques en enquête préliminaire ou de flagrance et les rendre applicables à la quasi-totalité des crimes et délits dans les mêmes conditions que les interceptions réalisées dans le cadre de l'information judiciaire. Le seuil retenu de trois ans d'emprisonnement encourus inclut la quasi-totalité de la masse des délits de droit commun, à l'exception notable des infractions routières, des dégradations légères et des délits d'outrage et de rébellion. et de rébellion. Le rapport rendu à la Chancellerie par Jacques Beaume et Franck Natali dans le cadre des chantiers de la justice avait estimé qu'il n'était pas souhaitable de retenir un seuil inférieur à cinq ans d'emprisonnement encourus, seuil déjà abusivement bas. tel alignement des conditions des interceptions en enquête préliminaire ou de flagrance sur le droit commun des interceptions téléphoniques réalisées dans le cadre de l'information judiciaire est une négation de leur caractère dérogatoire, qui est donc banalisé. Cela entraîne un recul net et injustifiable de la garantie des libertés individuelles.

Au demeurant, les garanties prévues lors de l'enquête sont équivalentes à celles qui sont prévues pour l'instruction, et les écoutes seront dans dans les deux cas autorisées par un magistrat du siège dont les fonctions sont spécialisées, c'est-à-dire soit le juge d'instruction, soit le juge il me semble qu'il fallait évoluer. En réalité, la seule différence justifiée de régime entre l'enquête et l'instruction pour les interceptions téléphoniques est maintenue dans le projet que je défends. Elle concerne la durée de ces écoutes, qui sera évidemment bien plus courte lors de l'enquête que de l'instruction.

et des dérogations à ces différences qui rendent nos textes absolument incompréhensibles. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu harmoniser les seuils à trois ans ; tout le reste n'est pas justifié.

ailleurs, le projet réduit la durée pendant laquelle la géolocalisation pourra être mise en oeuvre sur la seule autorisation du parquet. Je le rappelle, les parquetiers sont des magistrats,

un point d'histoire. Nous avons voté la première loi française sur les techniques de renseignement. Nous l'avons fait parce que les techniques ont progressé- elles sont de plus en plus intrusives -et parce que, dans le même temps, le terrorisme s'est à plusieurs reprises emparé de l'actualité, dans des conditions dont tout le monde sait à quel point elles ont été tragiques. La convergence de cette actualité douloureuse et de ces innovations technologiques nous a conduits à encadrer l'utilisation des techniques de renseignement, notamment pour la prévention du terrorisme et la détection des groupes organisés préparant des attentats terroristes. Les attentats terroristes s'étant répétés, nous avons estimé avec le gouvernement de l'époque qu'il serait sage de permettre au juge d'instruction et, en partie, au procureur de la République de disposer des moyens donnés à la police dans le cadre d'une activité de renseignement pour prévenir Nous avons donc voté un certain nombre de dispositions, les plus importantes figurant dans une loi du 3 juin 2016. Je dois le dire, le Sénat a été aux avant-postes pour que les moyens donnés à la police le soient aussi à la à la justice. Mais il s'agissait de terrorisme et de grande criminalité. Aujourd'hui, on nous propose de faire un saut considérable.

infractions punissables de trois ans d'emprisonnement serait assorti de garanties, et vous avez essayé de nous convaincre que ces garanties seraient suffisantes. Ces garanties consistent principalement en l'intervention du juge des libertés et de la détention. Il se trouve que nos rapporteurs ont très longuement discuté avec les représentants des juges des libertés et de la détention. ils en ont retiré la conviction absolue que ceux-ci ne seraient pas en mesure d'exercer un contrôle utile sur l'exercice par les procureurs des pouvoirs que vous voulez leur donner. Il ne suffit pas d'avoir inscrit dans la loi des garanties formelles pour qu'elles se traduisent par une protection suffisante

à l'efficacité de la lutte contre l'insécurité, est de faire en sorte que l'équilibre que vous jugez satisfaisant et que nous jugeons insuffisant soit rétabli à la faveur de nos travaux. C'est tout l'objet

pas de même nature que ceux de la grande criminalité ou du terrorisme. Par ailleurs, il s'agit de faire en sorte que les garanties que nous voulons ajouter à celles que vous avez déjà prévues s'appliquent

débat. La philosophie de la commission, des lois qui se rattache à une longue tradition de notre assemblée, est la suivante : oui à davantage de moyens pour lutter contre l'insécurité, mais avec des garanties réelles et dans certaines limites dignes de notre tradition républicaine en matière de liberté.

il convient de maintenir le seuil de peine encourue de trois ans pour les interceptions de communication réalisées lors d'une enquête de flagrance ou préliminaire, à la place de celui de cinq ans retenu par la commission. En effet, ces écoutes doivent pouvoir être réalisées lors d'enquêtes menées pour des infractions telles que la soustraction d'un mineur par un parent, des vols ou des abus de confiance portant sur des sommes très importantes, sans qu'il soit comme actuellement nécessaire d'ouvrir une information qui inutilement encombrera les cabinets des juges d'instruction.

Il convient enfin de supprimer les complexifications introduites par la commission des lois par rapport au droit actuel en matière de géolocalisation. Ces complexifications tendent, d'une part, à réduire la durée de la mesure autorisée par le juge

Or il ne s'agit pas ici de faire référence à des techniques qui seraient exclusivement utilisées pour des questions liées au terrorisme,

De la même manière, comment peut-on affirmer qu'il n'existe pas de garantie formelle, alors même que, au-delà du JLD, le contrôle du procureur sur les enquêteurs et sur leurs demandes de placement de

Comment peut-on dire qu'il n'y a pas de garantie, alors que l'article 39-3 du code de procédure pénale précise clairement que le procureur enquête « à charge et à décharge

Mme Esther Benbassa. Le présent article étend le recours à la géolocalisation et aux interceptions, par la voie des communications électroniques, aux enquêtes préliminaires et de flagrance sur les crimes et délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement, comme cela se pratique déjà en matière de criminalité et de délinquance organisées. Cette mesure est une véritable atteinte au principe d'échelle des peines l'on passe au seuil de trois ans, de nombreux délits vont entrer sous le coup de ces dispositions, qui ne relevaient auparavant que de mesures d'exception destinées au crime. Le parquet pourrait demander des perquisitions et des écoutes téléphoniques pour des méfaits qui ne donnaient pas lieu jusque-là Nous ne pouvons accepter la banalisation de mesures spéciales qui viennent régulièrement s'incorporer, ces dernières années, au droit commun. Cette intégration dans le droit général est d'autant plus inquiétante qu'elle aboutit à une atteinte d'une exceptionnelle gravité aux libertés fondamentales. Nous nous devons de dénoncer les dangers liés à l'utilisation massive et sans garde-fous des dispositifs relevant des renseignements. Le présent amendement tend donc à encadrer cette pratique en incorporant dans l'article 27 le fait que le matériel collecté- écoutes, données de géolocalisation, etc. -ne pourra être produit devant le juge des libertés et de la détention pour justifier rétroactivement de l'intérêt de cette mesure. Si ce procédé est utilisé, il doit être limité à un intérêt préalable à son recours.

sur les amendements n 133, 231 et 27.

Ce qui n'était pas nécessaire pour le terrorisme le serait désormais pour des délits de droit commun punis d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, soit la quasi-totalité des délits de droit commun Il ne semble pas raisonnable non plus de confier de telles techniques d'enquête au parquet, qui ne présente pas des garanties similaires à celles des juges du siège. Peut-on imaginer de prendre des mesures très attentatoires aux libertés sans aucun contrôle d'un juge du siège ?

S'il aurait pu présenter une garantie intéressante au texte du Gouvernement, cet amendement ne semble pas correspondre au texte de la commission, qui a supprimé toute possibilité de confirmation rétroactive par le juge des libertés et de la détention. Dans ce dernier texte, toute interception judiciaire doit être autorisée préalablement

nous nous abstiendrons sur cet article, tout en soulignant les efforts réalisés par la commission. de vote. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, ayant été rapporteur de projets de loi, par le passé, qui portaient sur le terrorisme, je me souviens que nous avons accru très sensiblement les moyens intrusifs qui ont été donnés à la puissance publique dans différents domaines, afin de lutter plus efficacement contre le terrorisme.

de procéder aux vérifications et aux contrôles nécessaires. Il est clair que le seuil retenu de trois ans d'emprisonnement, alors que la commission a proposé cinq ans, se traduira par une très forte extension du périmètre puisqu'il inclura la presque totalité des délits de droit commun, à l'exception des infractions routières, des dégradations légères et des délits d'outrage et de rébellion

partagée par un certain nombre de personnes qui oeuvrent dans le domaine de la justice. Nous voulons être très prudents sur ce sujet, car nous sommes très attachés aux libertés publiques.

de garantir totalement son statut. Cela n'exclut pas, bien sûr, qu'ici ou là il puisse prêter son concours à telle ou telle autre fonction ; mais il le fait volontairement et il ne peut en aucun cas être « déplacé »

limité à un usage destiné aux enquêtes en matière de criminalité et de délinquance organisées, soit pour des méfaits extrêmement graves classant cette mesure dans le régime d'exception. L'article initial du projet de loi était excessif, visant à généraliser cette mesure à toutes les enquêtes liées à un délit ou à un crime entraînant une peine d'emprisonnement. Cette extension paraissait dangereuse en ce sens qu'elle mettait fin au monopole de l'emploi de cette disposition par des services spécialisés, alors même qu'une telle technique d'enquête, équivalente à l'infiltration, ne saurait être efficace que si elle est réalisée par des personnels formés à la spécificité de la cybercriminalité et plus singulièrement aux techniques d'infiltration numérique. La commission des lois a assoupli le dispositif prévu par le texte en adoptant un amendement du corapporteur, ramenant l'extension de cette mesure aux infractions passibles d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement. Elle a également ajouté un contrôle accru des magistrats lorsqu'une enquête sous pseudonyme sera diligentée. Mes chers collègues, nous notons évidemment les améliorations et apports venus modifier l'article 28. Nous réprouvons simplement le recours à ce type d'enquête, qui porte atteinte au principe de la loyauté de la preuve. Voilà pourquoi le présent amendement vise à supprimer l'article 28.

Introduite en 2007 dans le but de constater des infractions de mise en péril des mineurs, notamment en lien avec la pédopornographie, la procédure d'enquête sous pseudonyme a, par la suite, été élargie à d'autres contentieux tels que ceux qui sont liés à l'environnement, à la santé publique, etc. Il résulte des réformes successives plusieurs dispositions éparses dans le code de procédure pénale, dont la rédaction n'est pas harmonisée, ce qui nuit à la lisibilité et à l'efficacité du dispositif.

maintenir le principe selon lequel l'autorisation du magistrat pour acquérir ou transmettre des contenus ou produits illicites peut être donnée par tout moyen. Le fait de prévoir une décision écrite et motivée du magistrat nous semble alourdir inutilement la procédure et ne va pas dans le sens de la simplification, laquelle est, je le rappelle, l'un des objets principaux du projet de loi que je nous ne souhaitons pas restreindre la procédure d'enquête sous pseudonyme aux délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement, pour les raisons suivantes. proposons à l'ensemble des délits punis d'une peine d'emprisonnement tire les conséquences du développement généralisé des services de communication au public en ligne, ainsi que de l'importance prise par ces services dans la vie économique de notre pays.

qui ne porte pas atteinte, contrairement aux autres techniques spéciales d'enquête- écoutes téléphoniques, géolocalisation, etc. -, au droit au respect de la vie privée, dès lors que les contenus mis sur internet l'ont été par les auteurs des infractions eux-mêmes. Enfin, et surtout, la restriction aux seules infractions punies d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement proposée par la commission des lois constituerait, je le répète, un recul par rapport au droit actuel dans des affaires pour lesquelles cette procédure est aujourd'hui possible. par exemple, aux affaires d'acquisition ou de consultation d'images pédopornographiques qui constituent un délit puni de deux ans d'emprisonnement.

le fait de prévoir l'autorisation du procureur de la République ; le rappel que l'incitation, la provocation ou le recours à ce stratagème pour commettre une infraction sont prohibés, afin qu'il ne soit pas porté atteinte au principe de la loyauté des preuves.

n° 29 rectifié. Le présent article tend à unifier le régime juridique applicable aux techniques spéciales d'enquête de sonorisation, de captation d'images, de recueil des données techniques de connexion et de captation de données informatiques. Dans sa version initiale, il ouvrait également la possibilité de recourir à ces techniques spéciales d'enquête pour les crimes, et pas seulement pour les seules infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées. Si la commission des lois est parvenue à revenir sur cette extension, l'article proposé par l'exécutif reste problématique, car il vise à incorporer dans le droit commun des dispositions qui, jusque-là, appartenaient au régime d'exception. Si le présent article entrait en vigueur, les officiers de police judiciaire pourraient utiliser un appareil ou un mécanisme permettant la détection de conversations à distance ou la captation de données informatiques. Alors même que notre assemblée a récemment légiféré sur la question des données personnelles, il semble préjudiciable que nous portions une telle atteinte aux libertés fondamentales et au respect de la vie privée. Pour cette raison, cet amendement vise à supprimer l'article 29. La

à tous les crimes, et non plus seulement aux seules infractions qui relèvent de la criminalité et de la délinquance organisées. Il nous semble en effet que la particulière gravité des infractions que le législateur qualifie de crimes, et qui sont punies d'au moins quinze de réclusion criminelle, justifie que ces techniques soient utilisées pour rechercher leurs auteurs, qu'il s'agisse par exemple d'assassinats, d'une série d'homicides, de viols ou d'enlèvements, notamment de mineurs. L'impossibilité actuelle de recourir à ces techniques dès les premières heures de l'enquête prive les enquêteurs de moyens permettant d'orienter efficacement les recherches, de privilégier ou d'écarter rapidement certaines hypothèses d'enquête.

ne s'effectue pas dans la durée puisqu'il s'agit de saisir un stock de données. Cette disposition opère également une confusion avec la captation de données informatiques qui peut, quant à elle, s'inscrire dans la durée, puisqu'il s'agit d'intercepter un flux de données.

aux biens, en particulier les vols en bande organisée. Cela constitue par ailleurs un recul par rapport au droit existant, qui prévoit déjà cette faculté.

explication de vote. Madame

est prise par un juge qui appréciera la nécessité de recourir à ces moyens. D'autre part, les éléments qui seront issus de la mise en place de ces techniques spéciales d'enquête pourront faire l'objet d'un recours en nullité lorsqu'ils seront soumis au débat contradictoire, pendant l'instruction

spéciales d'enquête, afin d'y apporter plus de lisibilité. Elle a également complété le dispositif par un ensemble de garanties bienvenues : limitation à vingt-quatre heures de la durée d'autorisation de la technique, très intrusive, de captation des données informatiques ; exigence d'une ordonnance écrite et motivée

; interdiction, à peine de nullité, que les opérations aient un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées par les autorisations ; interdiction de conserver des séquences relatives à la vie privée qui sont étrangères aux infractions visées dans des décisions autorisant la mesure ; suppression de la nécessité pour le juge d'instruction, lors des informations

En effet, des difficultés particulières se posent avec les langues rares. Les interprètes étant peu nombreux et généralement connus dans les « communautés », ils sont régulièrement l'objet de pressions et de menaces sur eux-mêmes ou leur famille. Cet amendement reprend une disposition qui avait déjà été adoptée par le Sénat lors de l'examen de la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la justice pénale, en janvier 2017. J'ose espérer que cette mesure sera adoptée de nouveau aujourd'hui. Quel

du moins telle que nous l'avons comprise, puisque l'interprète ne fait que traduire des propos émis par d'autres. La comparaison avec le témoin, pour lequel il existe la possibilité de déposer sous X, ne me semble pas opérante. Le témoin peut bénéficier d'une protection parce qu'il est susceptible d'apporter des éléments de preuve, ce qui n'est pas le cas de l'interprète. Par ailleurs, la possibilité pour le traducteur de ne pas déclarer son adresse est déjà prévue par le droit existant, qui n'exige pas cette mention en procédure,

pour son application, la commission des affaires économiques a émis un avis favorable, par 31 voix pour et 3 bulletins blancs, à la nomination de M. Bernard Doroszczuk aux fonctions de président de l'Autorité de sûreté nucléaire.